deux précisions. L'article 5 a pour objet de clarifier la répartition des compétences et des qualités de chefs de file des collectivités et de leurs groupements en matière de transition écologique. Nous avons besoin de clarification entre les différentes strates de collectivités territoriales pour la bonne lisibilité de l'ensemble des politiques publiques relatives à la lutte contre le changement climatique et à la protection de la biodiversité. C'est pourquoi il paraît nécessaire que leurs attributions et leur champ d'intervention soient inscrits de manière explicite dans le droit positif et que certains contenus de chefs de filât soient

La prévention de la production de déchets dont elles sont désignées les chefs de file est à la base de l'économie circulaire et vise à préserver les ressources- matières premières primaires et ressources naturelles.

constitue le cadre politique de référence pour l'action des régions en matière d'aides aux entreprises et à l'investissement immobilier, de soutien à l'innovation des entreprises et d'appui à l'attractivité du territoire régional. L'évolution de nos modes de consommation, la prise de conscience des enjeux de la préservation de l'environnement, du développement durable et de la lutte contre le changement climatique incitent à encourager et à soutenir les initiatives en matière d'économie circulaire. Pour ce faire, il est nécessaire que la stratégie régionale, dans le domaine économique, l'intègre pleinement et y consacre un volet de son schéma. Les deux amendements

permettent de penser qu'une rupture vis-à-vis de notre modèle de production, de consommation ou, plus généralement, de surconsommation, est non seulement souhaitable, mais possible. Ainsi, le déploiement d'une économie circulaire doit être organisé par une gouvernance locale adaptée aux besoins, adaptée aux besoins, aux spécificités d'un territoire et de ses habitants. Activités économiques locales, présence de ressources et de débouchés, caractéristiques géologiques et climatiques, spécificités de production, seuils d'acceptation

L'accès à l'eau et à l'assainissement est une compétence propre aux collectivités qu'il importe de mettre en oeuvre, compte tenu notamment de la directive européenne 2020/2184 du 16 décembre 2020 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. Si les droits à l'eau et à l'assainissement sont déjà très largement mis en oeuvre en France, il existe encore plus de 300 000 personnes privées d'accès à l'eau et près d'un million de personnes pour qui l'eau est inabordable.

et instaurent une priorité en faveur de l'alimentation des personnes en eau potable.

janvier 2023. En l'état actuel du droit interne, aucun texte n'impose expressément à l'État et aux collectivités territoriales de prendre des mesures pour garantir l'accès à l'eau des groupes de personnes vulnérables et marginalisées. Dans le silence des textes, le juge administratif oblige les maires et les préfets au titre de leurs pouvoirs de police générale à créer des points d'eau pour les campements illicites, entre autres. Les mesures proposées ici créent de nouvelles obligations pour les collectivités, ainsi que l'ont rappelé les sénateurs

Si les droits à l'eau et à l'assainissement sont déjà très largement mis en oeuvre en France, il existe encore plus de 300 000 personnes sans accès à l'eau et près d'un million de personnes pour qui l'eau est inabordable. de nombreuses initiatives parlementaires ont été menées sur ce sujet, aussi bien par le groupe socialiste, depuis 2017, que par le groupe CRCE il y a quelques mois, elles n'ont jamais abouti, si bien qu'aucune solution durable n'est aujourd'hui apportée aux personnes qui se trouvent dans une situation de grande précarité.

Nous souhaitons également que les collectivités rendent publics les emplacements des points d'eau et des toilettes publiques. La plupart des personnes ont besoin d'avoir connaissance des infrastructures sanitaires.

la date limite de décision du report de transfert de compétence. Surtout, elle a accordé aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération la faculté de déléguer, par convention, tout ou partie des compétences eau et assainissement.

traiter consciencieusement le problème de l'alimentation en eau, tant pour les hommes que pour les animaux et l'agriculture, que par le partage des compétences. Les intercommunalités peuvent supporter à la fois le coût du fonctionnement

? Madame la ministre, vous venez de rappeler que l'eau, plus encore que l'assainissement, est un sujet qui revient chaque fois que nous débattons dans cet hémicycle

À y regarder de près, on constate que, depuis le processus d'intercommunalisation de la gestion de l'eau et de l'assainissement,

Vous voulez absolument nous imposer ce qui serait bien pour nous, parce que vous pensez savoir mieux que nous ce dont nous avons besoin ; vous voulez faire le bien de ceux qui ne sont pas

Après 2026, on risque d'assister à deux phénomènes négatifs : l'effacement de la gestion par les communes

un contrôle citoyen du pacte de délégation de pouvoir établi au moment des élections. Cela demeure fondamental dans un siècle où la question de la

concerné. Madame la ministre, heureusement qu'il y a des interconnexions en matière d'eau, mais vous savez comme moi qu'il existe des communes en interconnexion avec une gestion communale de l'eau.

n° 340 rectifié . Cet amendement vise à permettre la délimitation des zonages des eaux pluviales avant 2026, sur la base d'un diagnostic tenant compte des effets du changement climatique. Les eaux pluviales, du fait de leur ruissellement sur des surfaces imperméabilisées souvent souillées, constituent une source de pollution importante pour les milieux aquatiques. Les états des lieux réalisés dans le cadre de l'élaboration des schémas directeurs de gestion des eaux pluviales mettent en évidence la contribution importante des eaux pluviales à la Les communes et établissements publics de coopération intercommunale en charge d'un service public de gestion des eaux pluviales délimitent, en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les zones où des mesures spécifiques doivent être prises pour la gestion des eaux pluviales, au regard d'enjeux quantitatifs et qualitatifs. Elles doivent également maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages et équipements rattachés à ce service. Le changement climatique contribue à accroître les tensions qui s'exercent sur la ressource en eau. Des pénuries sont constatées et touchent désormais l'ensemble du territoire. Des phénomènes de pluies intenses et les inondations qui en découlent sont également constatés de plus en plus fréquemment. Dans ce contexte, il paraît nécessaire que l'ensemble du territoire national soit, dans les meilleurs délais, couvert par des zonages d'eaux pluviales afin que soient définies et appliquées les mesures nécessaires pour répondre, au regard des spécificités de chaque territoire,

augmenter excessivement les contraintes pesant sur les collectivités territoriales en la matière. Au surplus, la définition du diagnostic tenant compte des effets du changement climatique semble assez lacunaire et crée un risque contentieux. C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.

? Madame la sénatrice, il va de soi qu'un tel assouplissement ne pouvait être accordé qu'aux syndicats d'eau potable et d'assainissement existant à la date de la publication de la loi

Faute de pouvoir se conformer à ces règles, un grand nombre de communes rurales de ces départements sont contraintes de refuser toute demande de permis de construire sur leur territoire.

Ces missions peuvent être financées par la taxe dite Gemapi, prévue à l'article 1530 du code général des impôts. En vertu de l'article L. 213-12 du code de l'environnement, les collectivités territoriales peuvent s'appuyer

Ce prélèvement constituant une taxe additionnelle aux taxes foncières, son produit est fonction du nombre de contribuables que comprend l'EPCI, alors que le linéaire de digues à prendre en charge n'est pas lié à la démographie.

qu'elles soient sonores ou d'encerclement, sans parler de la question de l'artificialisation des sols et des problèmes de démantèlement à venir.

ayant une sensibilité écologique forte que, pour des raisons différentes, les régions sont hostiles non pas aux éoliennes en tant que telles, mais aux éoliennes mal réparties ou trop nombreuses. Il se trouve qu'à titre personnel

Il s'agit de renforcer le pouvoir des maires en cas de projets d'installation d'infrastructures de transport par câbles en milieu urbain sur le territoire de leur commune. En effet, bien que ces infrastructures poursuivent une mission de transport en commun, elles revêtent une dimension urbanistique et esthétique qui a de

est de constater que l'implantation d'éoliennes pose la question majeure de l'acceptabilité. Il convient donc d'établir des concertations en amont, en impliquant les populations locales représentées par l'ensemble des communautés de communes du territoire, pas seulement les maires. Les réflexions locales pour une cartographie des implantations d'éoliennes doivent aboutir à un développement harmonieux, accepté par les populations et les territoires, dans un échange de démocratie locale.

de récupérer des portions de routes nationales, l'ensemble des collectivités- régions, départements, métropoles -doivent pouvoir bénéficier d'une information claire sur les contraintes liées à de tels ouvrages. Aussi, cet amendement vise à demander au Gouvernement la publication d'un rapport détaillé, notamment sur les coûts liés à ces routes

de concertation. Nous en avons longuement discuté avec les collectivités concernées et avec les rapporteurs. Il nous semble utile d'inscrire dans la loi l'ensemble de ces concertations, afin que les transferts et mises à disposition de routes,

été voté, un nouveau cycle de concertations avec les collectivités intéressées, sur la base de la carte des routes décentralisables que nous vous avons communiquée.

chaque sénateur, peut prendre connaissance de l'ensemble du dossier. Le processus évoluera en concertation avec les départements et les régions.

Cet amendement vise à compléter l'alinéa 2, pour que des informations qualitatives sur les flux de circulation et les possibilités de développement des alternatives à la voiture individuelle, sur les routes ou portions de route transférables, puissent être transmises aux collectivités territoriales. en commission, les rapporteurs ont introduit une disposition prévoyant une communication par les préfets aux collectivités qui en font la demande de toutes les informations permettant le transfert d'une portion de voie, autoroute ou route relevant du domaine public non concédé. Nous sommes favorables à une telle disposition, qui permet aux collectivités concernées de mieux apprécier les routes susceptibles de faire l'objet d'un transfert, avant même d'en faire la demande. Cependant, nous craignons que seules les informations techniques, certes nécessaires, ne soient transmises, alors que d'autres informations tout aussi importantes à nos yeux devraient également l'être. En effet, à l'heure de la nécessaire transition écologique, les collectivités ont un rôle majeur à jouer dans le développement des mobilités alternatives. Elles doivent donc avoir accès à l'ensemble des informations leur permettant d'assurer ce développement,

Les autoroutes représentent un enjeu particulier pour l'intérêt national, en matière de défense, de gestion de crise de garantie des flux économiques. Il est donc indispensable qu'elles restent aménagées de telle sorte que les convois exceptionnels pour alimenter les chantiers, par exemple les convois militaires, puissent continuer d'y passer. Il est également indispensable de s'assurer que les aménagements que la collectivité pourrait y faire ne dégraderaient pas l'accessibilité de certaines communes. Par conséquent, la décision de déclasser une voie de son statut autoroutier doit revenir à l'État, après avis de la collectivité propriétaire. Il est donc proposé de rétablir la rédaction initiale. M. Didier Marie. Sur l'initiative de ses rapporteurs, la commission des lois a confié aux collectivités territoriales et groupements propriétaires d'autoroutes ou de portions d'autoroutes la possibilité de déclasser le statut autoroutier de ces voies, après avis conforme du préfet coordonnateur des itinéraires routiers. Cette disposition nous semble poser des difficultés quant à la cohérence des itinéraires routiers et en matière de sécurité routière. Certes, il est prévu que cette faculté de déclassement ne peut être mise en oeuvre qu'après avis conforme du préfet coordonnateur. Cependant, quel serait le bénéfice pour les collectivités, si, en définitive, c'est le représentant de l'État qui décide ? Pour ces raisons, nous proposons de maintenir le droit en vigueur, qui prévoit que le déclassement du statut autoroutier est prononcé par décret, après avis de la collectivité propriétaire.

utilisés à la date du transfert exclusivement pour l'aménagement, l'entretien, l'exploitation ou la gestion des routes transférées. En effet, ces biens étant attachés à ces usages,

Les biens utilisés pour l'exercice d'une compétence transférée aux collectivités territoriales sont en principe mis à disposition des collectivités bénéficiaires de ce transfert de compétences. est le régime qui a été suivi pour l'application du transfert de certaines routes nationales aux départements, prévu par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Dans un souci de simplification, cet amendement tend à céder aux départements la propriété des biens mis à leur disposition pour leur permettre de gérer ou d'exploiter les routes qui leur ont été transférées en application de la loi. C'est d'ailleurs la solution qui a été retenue pour les routes qui seront transférées au titre de l'article 6 de ce projet de loi. En première analyse, le Gouvernement est donc favorable à la finalité que vise cet amendement. Toutefois, il préfère disposer d'un délai pour préciser la rédaction et, si nécessaire, les modalités de ce transfert de propriété.

les charges liées à ces emplois feront l'objet d'une compensation financière aux collectivités bénéficiaires du transfert. L'article 6 prévoit la possibilité que des autoroutes soient transférées en pleine propriété aux départements et aux métropoles, tout en conservant leur statut autoroutier.

des transports exceptionnels, des convois et des transports militaires et la desserte économique du territoire national, l'article prévoit, d'une part, que le préfet conservera le pouvoir de police sur ces autoroutes,

les portions de voies dans lesquelles le préfet exerce seul le pouvoir de police, ainsi que les cas dans lesquels son avis préalable sur les principales modifications apportées aux caractéristiques techniques des voies est requis.

Lorsque l'ouvrage est géré en régie, le péage ne peut assurer que la couverture totale ou partielle des dépenses de toute nature liées à la construction. En revanche, lorsque l'ouvrage est géré sous forme de délégation de service public,

et l'exploitation de cet ouvrage, lorsqu'il répond aux caractéristiques définies par le code de la voirie routière, indépendamment du mode de gestion choisi, c'est-à-dire concession ou régie. Le Gouvernement n'a pas de raison de s'opposer à cet amendement. Par conséquent, il s'en remet à la sagesse

Cette disposition a en effet de quoi interroger quant à la lisibilité des compétences des collectivités en matière de voirie routière. Les départements sont reconnus pour l'exploitation de leur domaine routier, alors que les régions ne disposent pas de telles compétences. Par ailleurs, le texte prévoit que les modalités de compensation seront fixées par convention entre l'État et chaque région concernée, mais en faisant référence aux règles d'évaluation favorables retenues pour les transferts définitifs. Ces règles consistent à prendre en compte la moyenne les coûts historiques constatés, en matière de dépenses de fonctionnement et d'investissement, sur une période pluriannuelle. Le Conseil d'État indique que ces dispositions relatives à la compensation des transferts de compétences définitifs, en ce qu'elles attribuent notamment des ressources fiscales pérennes aux collectivités concernées, ne sont pas adaptées à un dispositif expérimental. Pour toutes ces raisons, nous souhaitons supprimer cet article.

doivent être une raison suffisante pour que les régions participent financièrement et s'impliquent. En revanche, acter la possibilité pour les régions d'être autorités de gestion de routes nationales, et même d'autoroutes non concédées, serait une erreur. En effet, cela reviendrait à reproduire des transferts de compétences irréfléchis, comme nous en avons connus,

s'est constamment détourné des appels incessants lancés par les élus de ce département. J'ai cru comprendre que cette route nationale faisait partie des itinéraires qui avaient vocation à être transférés.

Il est proposé de donner aux régions la possibilité d'expérimenter une redevance pour les poids lourds utilisant le réseau routier national, exception faite des autoroutes et routes nationales à péage. C'est une mesure de cohérence avec l'article 7 de ce projet de loi qui permet aux régions, à titre expérimental, de gérer et d'aménager les autoroutes, routes et portions de voies non concédées relevant du domaine public routier national situées sur leur territoire. Le transport de marchandises routier représente un bilan carbone problématique. Il occasionne aussi, sur les axes qu'il emprunte, de nombreuses difficultés tant pour les pouvoirs publics que pour les autres usagers, notamment la saturation des voies et leur dégradation rapide. Ce dernier phénomène constitue une véritable problématique pour les finances publiques, alors même que l'État et les collectivités connaissent les plus grandes difficultés à entretenir le réseau existant. Une telle ressource permettrait de résoudre en partie cette difficulté. De nombreux pays étrangers, notamment les voisins directs de la France, ont déjà instauré des écotaxes, occasionnant ainsi un report du trafic des camions étrangers sur les axes routiers français, surtout lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à péage. Afin d'anticiper les mécanismes de déport consécutifs à l'instauration de taxes sur des portions seules de territoires, sans cohérence avec l'ensemble du réseau routier régional, il est proposé qu'au sein d'une même région une taxe sur les poids lourds ne puisse être adoptée sans l'avis conforme des autres départements de la région. Cette disposition s'applique quels que soient les éventuels transferts de compétences du réseau routier national.

qui vise à bien articuler et à harmoniser les compétences entre la région Grand Est et la Collectivité européenne d'Alsace, laquelle mettra en place une écotaxe d'ici à 2024. J'y insiste, il s'agit non pas de s'opposer à ce qu'une écotaxe similaire puisse être mise en place dans d'autres territoires, mais bien de préserver la pleine souveraineté de la compétence qui a été attribuée à la CEA depuis 2019. Les deux

le principe pollueur-payeur. Il s'agit d'agir avec une plus grande cohérence et une vision d'ensemble prenant en compte les grands réseaux routiers européens, en permettant à la région Grand Est de mettre en place

Il s'agit de préciser que la CEA garde la pleine souveraineté pour l'instauration d'une écotaxe sur son domaine public et, surtout, d'éviter que les usagers des autoroutes alsaciennes soient redevables de deux taxes du seul fait de l'utilisation de ces voies.

de la protection de l'environnement, dite loi Barnier, interdit les constructions ou installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations, au sens du code de la voirie routière, ou de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation. Ce transfert des routes donne l'occasion de renforcer les corridors écologiques et de mieux protéger les sols. Ces zones inconstructibles sont souvent sous-utilisées aujourd'hui. Elles pourraient pourtant représenter un véritable levier d'action pour devenir des dépendances vertes. vertes. Cet amendement vise notamment à recycler les friches présentes dans ces zones inconstructibles, pour renaturer les sols et contribuer à la lutte contre leur artificialisation. Ces espaces annexes pourraient ainsi être mieux valorisés ou renaturés, afin de les rendre favorables à la biodiversité et de participer à la résilience des territoires. De plus, cela répond à un objectif de sécurité routière et de développement des services écosystémiques, dans la mesure où le fait de rendre les sols fonctionnels permet de lutter, en cas d'intempérie, contre l'inondation des routes- sans parler des avantages en termes de captation de carbone. Ce serait tout bénéfice, en somme

M. Didier Marie. Pour faire face aux conséquences de l'épidémie de covid-19, de nombreux maires ont pris des arrêtés de police permettant des aménagements en faveur des cyclistes, des engins de déplacement personnel et des piétons, dans le but, d'une part, de limiter les émissions de polluants atmosphériques nuisant à la qualité de l'air, d'autre part, d'assurer la sécurité de la circulation des usagers dans un contexte où la croissance du trafic cycliste était de nature à accroître la congestion et les risques d'accidents. L'augmentation significative du nombre de cycles est documentée. La pérennisation de ces dispositifs, qui s'inscrit en cohérence avec les engagements de la France à limiter ses émissions de CO2 dans le cadre de l'accord de Paris et à diminuer ses émissions de polluants atmosphériques, conformément aux directives européennes sur la qualité de l'air et à l'injonction du Conseil d'État du mois de juillet 2020, nécessite dans certains cas la mise en oeuvre de procédures de concertation ou d'évaluation lourdes, au titre des dispositions des codes de l'environnement, de l'urbanisme et du patrimoine. Cet amendement vise à permettre le maintien des dispositifs de type « coronapistes » pendant la durée des procédures de concertation et d'évaluation environnementale. L'amendement

Nous pourrons alors voir, à l'issue de cette crise sanitaire, si la pratique du vélo continue sa progression au sein de la société. L'urgence climatique, le besoin de mieux vivre et l'activité physique sont des enjeux essentiels pour la population. Cet amendement vise à les faire reconnaître dans la loi. Quel est l'avis de

Comme quoi, on en apprend tous les jours ! Ces amendements visent à sécuriser juridiquement le maintien en place des pistes cyclables aménagées dans le contexte de crise sanitaire.

Le périmètre de ce nouvel établissement doit en effet permettre de répondre aux enjeux de mobilité du bassin de vie lyonnais. C'est pourquoi la région, du fait de ses compétences, y est intégrée au titre des services de mobilité qu'elle opère dans ce bassin et de sa qualité de chef de file des mobilités.

à due concurrence des services régionaux interurbains et scolaires, qui seront confiés au nouvel établissement. En tout état de cause, la suppression proposée remettrait en cause l'ordonnance récente et nécessiterait d'habiliter à nouveau le Gouvernement. Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable

en lien avec les collectivités, la métropole, le Sytral ou le pôle métropolitain, si elle souhaite, ou non, gérer la compétence transport sur son périmètre. Ce n'est pas à l'État de définir la composition de ce type de syndicat ! Madame la ministre, vous avez une vision des territoires et de la libre administration des collectivités qui ne va pas dans le sens du respect des élus locaux.